Monsieur le président, La séance est reprise. Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la gestion de la crise sanitaire. Dans la discussion de l'article 1, nous en sommes parvenus à l'examen de quarante-trois amendements

Cet amendement vise à exempter les clients des terrasses du passe sanitaire. En effet, les études montrent que les espaces extérieurs sont beaucoup moins contaminants. De plus, cela laisserait aux restaurateurs le temps de s'adapter à ces nouvelles mesures. à M. Guillaume Gontard. Cet amendement a pour objet d'encadrer le périmètre des activités soumises au passe sanitaire. Les activités en extérieur- terrasses, marchés de plein air, petite restauration dans les parcs et espaces naturels

Il est donc difficilement compréhensible que les plages des bases de loisirs y soient soumises, car elles ne présentent pas de facteur de risque supplémentaire. De même, par exemple, lors de la visite en voiture d'un parc animalier, le risque de contamination paraît inexistant. Ces activités de proximité sont souvent plébiscitées par les familles qui ne peuvent pas partir loin ; c'est la

M. Lucien Stanzione. En cohérence avec notre amendement déposé à l'alinéa 8 de l'article 1 de ce projet de loi, le présent amendement vise à exclure l'application du passe sanitaire aux activités se déroulant en plein air. En présentant cet amendement, nous ne minimisons pas l'impact de la propagation rapide du variant delta, car les activités de loisirs visées sont uniquement celles qui sont exercées en extérieur, où les risques de contamination sont plus faibles et où les règles sanitaires continuent à s'appliquer. Nous souhaitons également prendre en compte les conséquences d'une extension disproportionnée du passe sanitaire pour les professionnels du secteur autant que pour les Français qui profitent de ces activités de loisirs en plein air. L'amendement n° 116, présenté

l'on se presse pour aller visiter ce parc, qui permet de redécouvrir les traditions et la culture provençales, il est d'ores et déjà menacé par le passe sanitaire, qui démobilise les visiteurs potentiels. Pour la santé physique et psychique des Français et pour lutter contre les comorbidités, il faut permettre à nos concitoyens de garder un bon équilibre de vie, de s'aérer l'esprit et de faire du sport. L'expression « un esprit sain dans un corps sain » devrait, mes chers collègues, nous inspirer tous. Mais peut-être préférez-vous voir toutes les générations confondues se recroqueviller, pour ne pas dire s'abrutir, devant les écrans numériques ? En entendant les jeunes Français chanter le couplet « Liberté, liberté chérie », le 14 juillet, devant le Président de la République, j'ai ressenti de la fierté, mais j'avais aussi la gorge nouée. Le manque d'anticipation, l'incohérence et le dogmatisme ne doivent plus conduire à brader notre liberté. Les contradictions de notre société nous mènent à des extrémités frappantes : aujourd'hui, on aura de la compassion pour un animal sauvage retenu en cage. Je suis tout à fait favorable à ce que les animaux sauvages retrouvent la liberté, mais je suis surtout favorable à ce que les êtres humains puissent vivre en liberté ; or on leur accorde moins d'importance ! Mes chers collègues, je vous invite à peser à quel point la liberté d'aller et venir est fondamentale et à retirer les activités de loisirs de plein air du champ d'application du passe sanitaire en votant cet amendement.

La Défenseure des droits l'a rappelé dans un communiqué en date du 20 juillet dernier, « l'accès aux loisirs et à la culture est un droit proclamé par la Convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il ne s'agit pas d'un droit accessoire, mais bel et bien d'un droit fondamental pour le bon développement de l'enfant. » Cela a déjà été dit dans notre hémicycle, mais il ne me semble pas inutile de le rappeler. De plus, les avis scientifiques semblent diverger quant à l'équilibre entre bénéfice et risque pour les adolescents en plein développement qui, rappelons-le, ne subissent généralement pas, au moment où je parle- je reste prudente -de formes graves de la maladie. Cette crise sanitaire a déjà fait payer à la jeunesse, d'une manière générale, un lourd tribut. Il s'agit à présent de la préserver de cette vie

Nadia Sollogoub. Le présent amendement, déposé par ma collègue Sylvie Vermeillet, permet de laisser le libre choix de contrôle du passe sanitaire aux restaurateurs et cafetiers au sein de leur établissement, sans pour autant lever l'obligation de sa détention pour les clients. clients. Si le restaurateur ou cafetier souhaite sécuriser sa clientèle et s'il dispose du personnel pour le faire, il conserve un droit de contrôle et peut en informer ses clients. Cet amendement tend à prévoir l'organisation de contrôles de façon aléatoire au sein de ces établissements par les seuls agents disposant de l'autorité publique. Enfin, il vise à faire porter le risque de sanction et d'amende non plus sur les restaurateurs et cafetiers, mais sur les usagers, si ceux-ci ne respectent pas l'obligation de détention d'un passe sanitaire.

28 rectifié. Le présent article élargit les activités concernées par le passe sanitaire en incluant, par exemple, les activités de loisirs, les activités de restauration ou encore les foires et salons professionnels.

tandis que les protocoles sanitaires renforcés permettent de concilier l'activité de restauration et la protection sanitaire de la population. La parole

démontrant que les restaurants ou les bars seraient des lieux de contamination et des clusters en puissance. Ensuite, en pratique, les employés de ces établissements auront toutes les peines du monde à exercer leur métier, déjà éprouvant, à vérifier les passes sanitaires de chacun et à faire face aux clients récalcitrants. En outre, ces contraintes vont nécessairement conduire à un tarissement de la fréquentation de ces lieux et imposeront un énième coup d'arrêt à cette profession, déjà si durement touchée par la crise. Enfin, parce que les forces de l'ordre ne pourront pas toujours se rendre sur place aussitôt, les situations dégénéreront. Il est donc nécessaire de supprimer cet alinéa 10, dont la mise en pratique restera vaine.

Le passe sanitaire ne sera jamais un droit d'accès qui différencie les Français. Il ne saurait être obligatoire pour accéder aux lieux de la vie de tous les jours comme les restaurants, théâtres et cinémas, ou pour aller chez des amis. En ne respectant pas cet engagement, il perd un peu plus la confiance des Français. Avec le passe sanitaire imposé aux restaurateurs, la reprise économique paraît désormais fortement compromise. Pourtant, ceux-ci appliquent les restrictions et les protocoles sanitaires depuis de nombreux mois, alors qu'aucune étude épidémiologique ne démontre que les cafés et les restaurants seraient des lieux de contaminations. Pourquoi, alors, sont-ils ainsi montrés du doigt ? Qu'ont-ils fait de pire qu'un métro bondé ? Un restaurant est-il plus contaminant qu'une cantine d'entreprise ? Après de longs mois de fermeture imposée, cette disposition va alourdir la note pour les restaurateurs, qui comptaient sur cette période estivale pour se refaire une santé économique. La baisse, ou plutôt l'effondrement, du tourisme les a sévèrement impactés et beaucoup d'entre eux notent une fuite de leurs clients à cause des campagnes publiques de dénigrement de ces lieux de convivialité à la française. Ceux dont les salariés ne seront pas vaccinés devront fermer,

Plutôt que de contrôler la racaille et les trafiquants de drogue, ces policiers vont être envoyés dans les cafés, les bars et les restaurants pour contrôler les honnêtes gens et, éventuellement, les verbaliser.

On a appris, hier, que le passe sanitaire avait déjà entraîné une baisse de 70 % du nombre d'entrées depuis une semaine dans les cinémas. Belle performance ! La filière demandait un plan d'aide publique pour s'en sortir ; c'est maintenant le jackpot pour Netflix, Amazon Prime Je ne sais pas si vous pourrez revenir en arrière, mais votre temps est écoulé.

à restreindre le champ d'application du passe sanitaire aux espaces intérieurs des bars et des restaurants et à exclure son usage pour les terrasses. En effet, le risque de propagation du virus est beaucoup moins élevé en extérieur. Il n'apparaît donc pas justifié qu'une disposition aussi contraignante que le passe sanitaire s'y applique. L'amendement

permettez au moins que les terrasses ne soient pas soumises au passe sanitaire. Cet allégement des contraintes se fera au bénéfice des clients et des professionnels, et donc des caisses de l'État pensez au moins à cela ! Une telle mesure de votre part est disproportionnée, car il n'y a pas de circulation spécialement accrue du virus en plein air. De plus, les terrasses de nos bars, cafés et restaurants sont devenues, depuis les tragiques attentats islamistes du Bataclan, un symbole français de résistance. C'est pourquoi je vous invite à légiférer en cohérence avec notre mode de vie et avec notre objectif de relance économique : laissons les terrasses hors des chaînes du passe sanitaire.

Les professionnels veillent à respecter les protocoles sanitaires, car il y va de la sécurité de leurs clients et de la survie de leur activité. Il ne paraît donc pas raisonnable de leur ajouter une mission de contrôle dont la mise en oeuvre est difficilement applicable et peu efficace. Il convient donc de vaut uniquement pour les espaces intérieurs. Gay. Les confinements, la fermeture des établissements scolaires, des parcs, des jardins, des lieux de loisirs et de culture, tout cela a eu un effet délétère sur les enfants et les adolescents de notre pays. De nombreuses De nombreuses études et rapports, dont celui de notre collègue Marie-George Buffet, députée de la Seine-Saint-Denis, nous ont alertés sur la santé mentale et physique de nos enfants et de nos adolescents, sur leur apprentissage, mais aussi sur leur niveau de vie. Selon Santé publique France, les mineurs qui ont ressenti davantage de détresse sont ceux qui sont issus des familles plus fragilisées. Ce sont encore eux qui vont subir de plein fouet les restrictions liées au passe sanitaire.

En effet, il apparaît inconcevable que le passe sanitaire soit requis dès l'entrée en vigueur de ce texte, alors même que le délai d'obtention dudit passe est d'environ six semaines. L'obligation de présentation du passe sanitaire dans les lieux mentionnés à l'article 1 doit donc être fixée au 1 septembre 2021. Les deux Levi, pour présenter l'amendement n° 37. Après les annonces du Président de la République le 12 juillet dernier, les Français se sont rués massivement vers les centres de vaccination pour prendre rendez-vous dans les meilleurs délais. Cette situation est bien le signe que nos concitoyens ont entendu le message du chef de l'État. En pratique, ce regain se traduit par un allongement considérable des délais de vaccination. Désormais, une large partie de la population peine à obtenir une première dose de vaccin rapidement et il lui est encore plus difficile d'obtenir la seconde avant la date du 30 août 2021. C'est pourquoi la date du 1 octobre semble être plus appropriée pour tenir compte de ces contraintes organisationnelles.

l'amendement n° 92. Cet amendement de Mme Annick Billon vise à repousser de quelques jours le délai de mise en place du passe sanitaire dans les lieux recevant du public. Actuellement, 42,5 % des Français sont vaccinés, ce qui n'est pas suffisant pour atteindre l'immunité collective. Eu égard à l'élan des prises de rendez-vous de ces derniers jours, les primo-vaccinés se trouveraient, par voie de conséquence, exclus de certains lieux. Loin de tomber dans la précipitation gouvernementale de ces derniers jours, les auteurs de cet amendement entendent ne pas stigmatiser les citoyens, mais les convaincre de se faire vacciner. De plus, des inquiétudes remontent des exploitants de parcs de loisirs, de parcs animaliers et de parcs à thèmes, qui, loin de refuser la politique sanitaire, critiquent néanmoins l'impact de la mise en place précipitée du passe sur leur clientèle estivale. un décalage de l'entrée en vigueur de ce dispositif au 15 septembre permettrait de préserver la saison estivale et, par la même occasion, de protéger leurs marges financières, amoindries par les confinements successifs. Enfin, repousser la date d'entrée en vigueur de ce passe de quelques jours n'aurait aucun impact sur la campagne vaccinale.

visés par l'article 1 du projet de loi. Le délai actuellement envisagé est trop restreint pour permettre aux personnels intéressés de se faire vacciner dans les temps et de satisfaire ainsi à l'obligation requise. Certes, la vaccination n'est pas obligatoire, puisque vous ne l'avez pas souhaité, mais les personnels seront conduits à y recourir pour éviter de produire systématiquement

Le passe sanitaire que vous nous imposez doit être limité dans le temps et dans l'espace selon ce critère de gravité « avérée », qui se fonde sur l'incidence locale,

l'autoritarisme sanitaire. Oui, nous vivons une période d'exception. Non, les masques et les restrictions ne sont pas la norme et ne devront jamais le devenir ! Le masque ne devra pas devenir obligatoire à la moindre épidémie de grippe et la vaccination ne devra pas être imposée à tous au premier virus venu.

à qui Richard Ferrand, grand macroniste devant l'Éternel, refuse d'imposer le passe sanitaire sous prétexte que ce serait anticonstitutionnel. Il a raison ! On peut donc enfermer le pays pendant des mois, contrôler l'identité des gens qui se rendent au restaurant ; mais pour ce qui d'imposer aux députés ce

que vous vous moquez d'eux. Contre les abus de pouvoir répétés, inquiétants et dangereux, je vous demande de voter cet amendement de bon sens. S'il n'y a plus de virus, il faut lever les restrictions et supprimer les atteintes aux libertés. L'amendement n°

De ce fait, les adolescents de 12 à 18 ans disposent d'un accès à la vaccination plus restreint que le reste de la population, d'autant que seul le vaccin Pfizer est autorisé dans cette tranche d'âge et que la vaccination des mineurs de plus de 12 ans ne peut intervenir que dans des centres C'est pour toutes ces raisons, et notamment la première, que nous proposons de supprimer le passe sanitaire pour les mineurs, ce qui n'empêchera pas les pouvoirs publics d'encourager, après consensus scientifique, la vaccination pour les enfants de plus de 12 ans. Cet amendement s'appuie sur les avis du Comité consultatif national d'éthique, de la CNIL, de la Défenseure des droits et de très nombreux professionnels de santé de l'enfant.

Ce dispositif ne saurait en effet être pérennisé, sous peine de constituer une grave atteinte à la liberté d'aller et venir de nos concitoyens. Or le Gouvernement n'offre aucune garantie sur le caractère temporaire de ces justificatifs.

instruction. Beaucoup d'amendements recouvrent les mêmes problématiques. Ce qui est très intéressant pour notre débat, c'est que ces amendements proviennent de tous les groupes et qu'ils vont dans la même direction.

voire des grands-parents et, d'autre part, par les responsables de lieux d'accueil de jeunes. Nos jeunes ont un grand besoin de liberté après des mois et des mois d'une vie sous forte contrainte, et c'est un véritable crève-coeur que de devoir exercer une forme de surveillance sanitaire. Cependant, mes chers collègues, je me suis senti obligé d'analyser les faits scientifiques, les expérimentations, les études qui ont été produites. Or ces études sont convergentes : les jeunes âgés de 12 à 18 ans sont aussi contaminants, voire davantage que les adultes. Un très grand nombre d'études venant de plusieurs pays attestent de cette réalité. La Haute Autorité de santé (HAS) l'a confirmé de la manière la plus nette : ce n'est pas une hypothèse,

Mes chers collègues, tous les amendements ayant trait aux mineurs doivent aussi s'inscrire dans un contexte qui est celui du texte que nous avons adopté en commission. Or ce texte prévoit bien que l'on

Pour un certain nombre de restaurateurs et de gestionnaires de parcs d'attractions- j'y reviendrai -, établir une distinction entre l'extérieur et l'intérieur serait en réalité bien plus complexe à mettre en oeuvre

explication de vote. En ce qui me concerne, je suivrai l'avis de la commission des lois. Je vous demande surtout de bien réfléchir à certaines données importantes faciliter d'une façon ou d'une autre le transfert ou le voyage du virus d'une personne à une autre conduit obligatoirement, à un moment ou à un autre, à la mise en

la position du rapporteur : nous ne sommes plus dans un processus législatif tel que celui que vous nous aviez pu nous présenter, monsieur le de nouveau dans un dispositif de sécurité sanitaire généralisé. Il faut que le Gouvernement le reconnaisse et assume cette

prises pendant des mois ... Accepter le passe sanitaire dans les conditions que l'on veut nous imposer aujourd'hui, notamment en extérieur et dans les petits sites, c'est accepter l'idée que, depuis des mois, on nous raconte des carabistouilles

autant de cohérence que vous avez pu dans un texte qui, parfois, en manque. Mais, chaque fois que l'on souligne les failles du dispositif ou des contradictions telles que « oui au métro, non à la terrasse », cela affaiblit

Je souhaiterais particulièrement revenir sur l'exigence du passe pour les jeunes âgés de 12 à 18 ans. Hasard ou coïncidence, on peut tout de même remarquer que le passe sanitaire est exigé pour la majorité des lieux dont sont friands nos jeunes : les bars, les discothèques, les parcs d'attractions, les cinémas Je soutiendrai donc les amendements de Loïc Hervé et Henri Leroy, qui tendent à élever la limite d'âge à 18 ans. Dans notre pays où le principe de précaution est servi à toutes les sauces et sur tous les sujets,

Nous savions que le Gouvernement en avait été touché sévèrement et, manifestement, il semble que la commission des lois du Sénat est elle aussi atteinte. Peut-être Peut-être est-ce parce qu'il n'y a plus de distanciation physique que la distanciation politique se réduit ... Notre collègue Philippe Bas a justifié son rejet

: ce n'est ni au Gouvernement ni à la loi d'imposer ; c'est aux parents de prendre leurs responsabilités. Je ne connais pas de parents qui ne soient pas soucieux de la santé de leur enfant, qui ne se préoccupent pas de la contamination dont il pourrait être à l'origine. Les parents, l'autorité parentale, cela existe

À leur manière, ils m'ont expliqué qu'ils avaient du mal à faire respecter ne serait-ce que les règles de distanciation et de maintien du masque. C'est compliqué, et je sais que,

est à M. le rapporteur. À tous ceux d'entre nous qui plaident pour la cohérence, je veux dire que c'est aussi mon combat.

qualifierai d'« amendements terrasses », je crois réellement que les arguments scientifiques portés à notre connaissance sont absolument imparables. Manger et boire sont les moments où les risques de contamination sont les plus forts ; manger et boire dehors, dans la promiscuité, dans la proximité, est devenu aussi dangereux

ne perforez pas le dispositif du passe sanitaire, dont vous venez de voter le principe. J'en viens à la question des mineurs. Je crois que nous sommes en train de nous prononcer sur un malentendu, et je voudrais vérifier que ce n'est pas le cas. La règle, mes chers collègues, ce n'est pas que les mineurs vont être empêchés d'accéder, dès le vote de la loi, aux centres de loisirs, aux restaurants, aux cafés, aux théâtres, aux cinémas, aux lieux de culture, aux centres sportifs. C'est tout le contraire

Jeunes gens, je vous en supplie, soyez prudents ! Vous êtes exonérés de cette obligation pendant toute la période des vacances. Ne commettez pas d'imprudences

qui allez décider. Faites-le en votre âme et conscience. Je sais que vous avez tous, comme j'essaie de l'avoir aussi, un esprit de responsabilité et que vous cherchez le bon équilibre entre des mesures de protection sanitaire de la population, qui s'imposent compte tenu de la gravité de l'épidémie, et le respect d'un certain nombre de droits et de libertés fondamentales. Il faut dire, enfin, que si les règles changent, ce n'est pas par incohérence. C'est parce que le virus lui-même a changé et que la situation à laquelle nous sommes confrontés s'est modifiée elle aussi.

Cet amendement vise à simplifier le contrôle, donc l'organisation de l'activité des entreprises, et à alléger la responsabilité de l'employeur. Il est proposé d'instaurer un registre autodéclaratif, afin de permettre

nous tenons compte de situations qui sont parfois dramatiques et toujours complexes. Pour autant, face à ces situations-là, on ne va pas continuer à déconstruire

de vaccination établis par des organismes étrangers attestant la satisfaction aux critères requis par le justificatif de statut vaccinal ». Si je comprends bien, il faudra être « surdosé

amendement vise à adapter l'application du passe sanitaire dans les outre-mer pour tenir compte des caractéristiques particulières de ces territoires, avec concertation et en tenant compte du mode de vie des populations locales, ainsi que du système de santé lacunaire et de l'offre de service à mettre en place pour garantir le dépistage de tous les citoyens ne souhaitant pas recourir, pour l'heure, à la vaccination. En effet, en Guyane et dans les autres collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, le virus circule de manière différenciée au regard de ce qui a pu être observé sur le territoire hexagonal. Le taux de contamination augmente de manière régulière depuis l'ouverture aux frontières et la levée des motifs impérieux. Par exemple, selon les dernières statistiques de l'ARS, l'agence régionale de santé, de Guadeloupe, communiquées le 7 juillet 2021, quelque 112 nouveaux cas étaient recensés sur une semaine, incluant les touristes porteurs du virus, sur les 9 677 cas recensés quotidiennement sur le territoire national. territoire national. Le taux de couverture vaccinale des populations guadeloupéenne- 25,78 % -, martiniquaise- 15,33 % -, mahoraise et réunionnaise- 31,6 % -est faible et révèle une réticence évidente, justifiant d'éviter toute forme nouvelle de crispation généralisée.

tenant compte des revendications portées par une vingtaine de collectifs citoyens et associations, afin de manifester leur désaccord vis-à-vis de l'extension du passe sanitaire, du maintien des motifs impérieux pour circuler sur le territoire régional et de la vaccination obligatoire des soignants. En outre, les personnes non vaccinées, soit 80 % de la population, ne seront pas en mesure d'accéder de manière facilitée aux lieux de dépistage, laissant craindre une privation des droits les plus élémentaires pendant une période non évaluée. Plus grave, les Ultramarins seront privés de l'accès à leurs proches hospitalisés pour les mêmes raisons, alors même que ces sociétés sont profondément structurées autour des valeurs familiales. Il apparaît dès lors que l'extension du passe sanitaire à toutes les activités visées par l'article 1, sans distinction, sans adaptation et sans considération des flux de rencontre à l'échelle d'une population locale, est disproportionnée et aura de fortes conséquences socioéconomiques. Monsieur le secrétaire d'État, il est urgent de prendre en considération les contraintes particulières des collectivités régies par les dispositions de l'article 73 de la Constitution dans une logique de différenciation, telle que le Président de la République l'a revendiquée pour les territoires français.

dois dire que j'ai l'habitude d'entendre ce genre de déclarations. D'ailleurs, monsieur le rapporteur, vous avez conduit une mission en Guyane il n'y a pas très longtemps

Nombreux sont ceux qui ont commencé leur schéma vaccinal, mais celui-ci sera incomplet au 1 août, et ils ne pourront donc pas bénéficier du passe sanitaire. Pour ceux qui n'ont pas encore débuté leur schéma vaccinal, mais qui souhaitent activement le faire, les délais de rendez-vous se sont fortement allongés depuis les annonces du Président de la République. Afin de ne

Cet amendement vise également à ne pas pénaliser nos concitoyens qui se sont déjà engagés dans un parcours vaccinal ou ceux qui souhaitent le faire sans avoir pu encore obtenir de rendez-vous. C'est la raison pour laquelle je vous invite, mes chers collègues, à voter cet amendement de bon sens pour nos concitoyens.

Je vous rappelle ce qu'il nous disait à l'époque : « StopCovid n'est pas une coquetterie technologique. C'est un outil sanitaire au service de la protection des Françaises Soit on fait tout pour éviter que l'épidémie reprenne, soit on choisit de priver les volontaires de cette protection et on accepte qu'il y ait des contaminations et des morts.

l'urgence de la situation sanitaire dans laquelle nous nous trouvons, tout en reconnaissant l'utilité, parmi d'autres

est dommage de se priver de l'outil qu'est le passe sanitaire. Je vous le redis : en l'état actuel des choses, au vu des votes

documents permettant d'obtenir un passe sanitaire valide le résultat d'un examen de sérologie concernant la covid-19 et concluant à un taux de présence d'anticorps suffisant ; le seuil serait fixé par un décret,

amendement, déposé par notre collègue Alexandra Borchio Fontimp, vise à appeler l'attention du Gouvernement sur la différence de traitement entre les plages déléguées dans le cadre d'une exploitation commerciale et les espaces publics du domaine public maritime.

Pour le Gouvernement, il semblerait que nos concitoyens puissent contracter le virus en s'installant sur les lots d'accueil touristique et balnéaire concédés à des délégataires, où le respect des règles sanitaires est scrupuleusement contrôlé par leurs En revanche, le virus s'arrêterait aux portes des plages publiques, sur lesquelles la distanciation sociale ne peut pourtant être appliquée ou son contrôle véritablement effectué, particulièrement en cette période estivale. Par ailleurs, à Antibes Juan-les-Pins, dans les Alpes-Maritimes, les plages concédées et, plus largement, les espaces naturels- sable, galets, ou encore rochers -aménagés pour le service public d'accueil touristique et balnéaire ne sont pas considérés comme des établissements recevant du public, des ERP, de type « plein air ». Ainsi, le projet de loi ne peut appliquer aux espaces naturels de plein air du domaine public maritime, délégués ou non, la même réglementation qu'à un établissement recevant du public. Cet amendement a donc pour objet d'appeler le Gouvernement à la vigilance et de l'inciter à remédier à cette situation totalement incompréhensible pour tous les professionnels d'un secteur déjà fortement affecté par deux saisons touristiques contrariées. En conclusion, monsieur le secrétaire

Alors que cette période estivale constitue une occasion de relance pour les bases de loisirs, après une année difficile, le risque attribué à la prolifération du variant delta contraint avec responsabilité à renforcer les restrictions sanitaires. cet amendement, je propose d'accorder un traitement adapté à l'industrie des bases de loisirs, déjà durement touchée par la crise, en lui accordant une marge de manoeuvre supplémentaire. L'état des connaissances permet aujourd'hui d'estimer que les attroupements extérieurs ne sont pas à l'origine de la grande majorité des contaminations ils ne représenteraient que 10 % environ de celles-ci. Par ailleurs, les courants d'air dispersent facilement les virus et les rayons ultraviolets participent à leur destruction. Enfin, l'obligation du passe sanitaire dans les bases de loisirs constitue pour les gérants d'établissements un effort logistique supplémentaire et accroît le risque de perte de clientèle, notamment vis-à-vis de ceux qui n'ont pas eu le temps de finaliser leur parcours vaccinal. La dispense des bases de loisirs de l'obligation du passe sanitaire nous paraît donc une mesure cohérente, compte tenu des risques évalués aujourd'hui. Quel est l'avis de la commission ? Comme pour mon cher collègue, je vous dirai : réjouissez-vous, grâce à un vote précédent du Sénat, point de passe sanitaire pour accéder aux pédalos

Noël. Cet amendement vise à reporter au 30 août l'application du passe sanitaire pour les encadrants, animateurs et directeurs d'accueils collectifs de mineurs, ou ACM, que sont les colonies de vacances, centres de loisirs et camps scouts. 2021, les mineurs sont exemptés de présenter un passe sanitaire. Grâce à cet aménagement, les mineurs pourront visiter des musées, accéder à des bases de loisirs et effectuer des visites culturelles dans le cadre de séjours de vacances. Cependant, cet aménagement permettant aux enfants et aux jeunes mineurs d'accéder à ces droits se trouve aussitôt remis en cause par le fait que les encadrants, animateurs et directeurs qui accompagnent ces mêmes enfants et jeunes doivent quant à eux présenter un passe sanitaire, à chaque sortie dans un musée, une base de loisirs, ou un lieu culturel, et même dans le cadre des déplacements de longue distance nécessaires pour se rendre sur le lieu du séjour. Les ACM doivent être vus comme un tout inséparable comprenant les mineurs accueillis, les animateurs et les directeurs, qui s'engagent auprès de ces enfants et de ces jeunes. Les animateurs et directeurs engagés pour l'été feront face à de grandes difficultés pratiques pour réaliser les tests PCR ou d'autres examens de dépistage réalisés moins de quarante-huit heures avant l'accès à l'établissement, au lieu ou à l'événement, surtout au milieu d'un séjour où tout est déjà préparé, cadré et finalisé. On peut aisément imaginer ces mêmes difficultés pour un séjour culturel, avec visites de musées et de lieux patrimoniaux, ou encore pour un séjour axé sur la visite de parcs d'attractions. En outre, pour tous les animateurs et directeurs qui ne sont pas encore vaccinés, il est impossible de présenter un schéma vaccinal complet avant quelques semaines. Ils sont donc contraints de réaliser chaque fois un test PCR, avec les complications pratiques précitées. Dès aujourd'hui, les acteurs des séjours de vacances et d'accueils de loisirs font part de démissions de directeurs et d'animateurs. Cela suscite de très grandes difficultés pour les organisateurs d'ACM, et ce dans un contexte de grande pénurie d'animateurs et de directeurs, encore aggravée par la situation sanitaire. C'est pourquoi nous avons déposé cet amendement, qui vise à aménager l'application des restrictions sanitaires, en les reportant au 30 août 2021 pour tous les animateurs et directeurs de colonies de vacances, centres de loisirs et camps scouts, dans la mesure où ces derniers agissent sur le temps de travail.

il me semble que, si nous avons accepté la possibilité que les mineurs se contaminent entre eux, puis aillent contaminer leur famille, leurs amis et les autres générations, on peut en revanche encore se soucier de les protéger contre les risques de contamination qui pourraient venir de leurs encadrants. C'est la raison pour laquelle je vous suggère, sur la pointe des pieds, avec beaucoup de précautions et sans vouloir vous forcer la main, mes chers collègues, de ne pas adopter ces amendements.

Par cet amendement, nous souhaitons exclure de l'élargissement du passe sanitaire les seules personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans les services et établissements de santé sociaux et médico-sociaux. Les personnes malades, les femmes enceintes, les personnes âgées, comme d'autres publics d'ailleurs, ne sauraient être privées de voir leur famille. Il est inutile de rappeler que l'isolement et la solitude des personnes âgées lors du premier confinement ont eu des conséquences très graves sur leur santé psychique. Il convient

Les résidents des maisons de retraite ont été victimes d'isolement et de déconsidération depuis un an et demi. Beaucoup en sont morts. De plus, les soignants seront encore les victimes de cette mesure, puisqu'ils devront affronter, à la place du Gouvernement, des situations particulièrement inhumaines. Cette orientation est insupportable. Cette vie que vous nous concoctez est un enfer. Rejetons donc cette inhumanité liberticide en supprimant cet alinéa. la Fédération hospitalière de France, qui regroupe plus de 1 000 hôpitaux et environ 3 800 établissements médico-sociaux, indique que cette mesure coûtera 60 millions d'euros par mois aux hôpitaux.

L'incapacité de milliers de Français à accompagner un parent dans ses derniers jours, le délaissement des personnes âgées privées de visites, l'explosion du mal-être, font malheureusement partie du bilan de la crise sanitaire.

Nous pouvions espérer que, dans cette situation, un droit de visite opposable aux patients, aux familles et aux accompagnants soit garanti. Or l'alinéa 12 prévoit l'inverse, puisque l'accès aux services et établissements de santé sociaux et médico-sociaux sera soumis à l'exigence d'un passe sanitaire pour les soins programmés, ainsi que pour les personnes qui accompagnent les patients. C'est donc une remise en cause du droit de visite des malades à l'hôpital, dans une situation déjà extrêmement dégradée de ce point de vue. Même en partageant l'objectif qui est visé par le passe sanitaire, et quand bien même nous le discutons, nous pensons que cette contrainte est disproportionnée et déshumanisante et qu'elle n'est pas acceptable dans cette situation. C'est pourquoi nous proposons la suppression de cet alinéa.

programmés. Ainsi, les patients se rendant à l'hôpital pour un autre motif qu'une urgence, notamment un rendez-vous prévu de longue date, devront présenter un passe sanitaire valide.

qui nous paraît prendre en compte l'ensemble des situations auxquelles ont été confrontées les personnes en grande fragilité. Le rapport de la Défenseure des droits du 4 mai dernier sur les droits fondamentaux des personnes âgées accueillies en Ehpad témoigne d'un nombre important d'établissements ayant fait l'objet de réclamations et où les visites n'ont été possibles qu'à une faible fréquence : visites hebdomadaires, parfois moins fréquentes encore, voire bimensuelles, limitées à trente ou quarante-cinq minutes, sur des plages horaires pouvant être imposées et, en tout état de cause, systématiquement limitées à un ou deux visiteurs. Plus encore, ce rapport mentionne que les aidants familiaux se rendant habituellement quotidiennement dans les Ehpad, notamment pour aider leurs proches à s'alimenter, n'ont guère obtenu de dérogations à ces limitations de visites. Il relate même des situations tragiquement ubuesques, telles que l'interruption brutale du repas en raison de la fin du temps de visite octroyé. Les résidents et leurs proches ont rapidement constaté que le rapport entre le nombre de créneaux de visites et le nombre de résidents limitait de fait les possibilités de visites, notamment en raison de l'insuffisance de personnels des établissements mobilisés pour organiser et surveiller le bon respect des gestes barrières. Pour les personnes d'ordinaire fortement entourées, notamment celles dont la famille est nombreuse, cela a conduit à étaler sur plusieurs mois les visites de leurs proches. Les conditions de visite ont été couramment décrites comme celles d'un « parloir » de personnes en détention, sous la surveillance d'un membre du personnel. Le respect des gestes barrières- port du masque, respect d'une distance d'au moins deux mètres et, parfois, présence d'une paroi en plexiglas -a rendu la communication impossible, notamment avec les personnes souffrant de malvoyance, de déficience auditive ou de pathologies dégénératives. Ces mesures sont inacceptables et indignes. Elles sont attentatoires aux droits et libertés fondamentaux et revêtent par là même un caractère disproportionné.

Premièrement, on ne peut pas exiger le passe sanitaire en cas d'urgence quand on accompagne quelqu'un ou quand on rend visite à quelqu'un. C'est la traduction qu'a donnée le Gouvernement à la demande de Bruno Retailleau, qui a proposé une loi à cet égard : si l'on doit rendre visite à un parent dans les derniers instants de sa vie, on entre dans ces cas d'urgence et on n'a pas à produire le passe sanitaire. C'est clair et net, mais je préférerais que M. le secrétaire d'État le confirme. Je le ferai ! Je sais que le Gouvernement l'a dit. Nous sommes absolument attachés à cette exigence humaine parmi les plus fondamentales au moment du grand passage, pour reprendre les termes mêmes utilisés par Bruno Retailleau dans son intervention en discussion générale.

soins sont programmés. C'est d'ailleurs l'occasion de rappeler que le passe sanitaire n'est pas une interdiction d'accès. C'est même exactement le contraire : c'est une permission d'accès ! En effet, il n'est pas difficile de se procurer le passe sanitaire si l'on a le temps d'anticiper

les personnes hospitalisées ou en maison de retraite. Il vous sera proposé tout à l'heure de voter l'obligation de vaccination pour les personnels. C'est une très lourde contrainte que, je pense,

de leurs auteurs, mais tout simplement parce qu'il me semble que les dispositions qui ont été adoptées en commission sont raisonnables et permettent de régler toutes les situations humaines que vous avez à l'esprit.

Dans le droit en vigueur, seuls les déplacements extrahexagonaux étaient concernés par la présentation de documents attestant de l'absence de contamination au virus. Le champ d'application de la mesure était précisément circonscrit. Tel n'est pas le cas de la notion de déplacement national de longue distance. Alors que la présente mesure prévue par le projet de loi risque de limiter considérablement la liberté d'aller et venir, même si elle n'est pas conditionnée par une obligation vaccinale et reste limitée dans le temps, on ne peut que regretter l'imprécision de la formulation retenue par le Gouvernement. Dans ce cas précis, l'intelligibilité de la loi fait défaut. Compte tenu de la couverture de transport différente selon les territoires et les modalités de transport- TGV ou TER -, qui ont une incidence directe sur le temps de déplacement, nous craignons un risque de rupture d'égalité entre citoyens. Il n'est pas acceptable de renvoyer toutes les conditions d'application de ce dispositif à un décret, en dépit de l'avis du Conseil d'État en ce sens.

pour Amsterdam, il faut avoir le fameux document européen ; en revanche, quand on prendrait l'avion pour Marseille-

la mesure. Le Sénat maintient les TER dans la liste des modalités de transport qui font l'objet d'une obligation de présentation de passe sanitaire, d'autant plus que le Gouvernement ne manquera pas de revenir à à sa rédaction. En effet, l'alinéa 13 étend le passe sanitaire aux longs trajets sur le territoire national par train, autocar ou avion. Nous ne reviendrons pas sur l'opportunité d'instaurer arrêterons sur les modalités pratiques d'application : manifestement, ce n'est pas si simple ! De manière particulière, les discussions à la SNCF sont vives : tous les trains ne seraient pas concernés. Seuls le seraient les TGV et les trains

la Défenseure des droits considère que « cette atteinte à la liberté d'aller et venir, envisagée de manière générale et sans information préalable délivrée suffisamment longtemps en amont, n'apparaît pas proportionnée à l'objectif de sauvegarder la santé publique qu'elle poursuit. » Enfin, la question du respect de cette mesure est encore assez floue. En effet, bien que les quelque 3 000 agents de contrôle soient déjà rompus, depuis le premier confinement, à la mise en place, dans des délais extrêmement courts, d'un dispositif de contrôle physique

je souhaite que le ministre réponde à une question qui nous a été souvent posée et qui concerne le transport maritime, notamment entre le continent et un certain nombre d'îles au large de la Bretagne ou de la Vendée. L'esprit du dispositif est que des passagers qui se côtoient sur une longue distance,

en cohérence l'obligation de présentation de ce passe à l'accès au Parlement et aux organes délibérants des collectivités territoriales. Afin que le dispositif proposé ne soit pas excessif au regard des modalités d'application retenues par ailleurs, il est précisé que cette obligation ne s'appliquerait que lorsque ces lieux rassemblent un nombre de personnes au moins égal à un seuil défini par décret. Le présent amendement vise bien évidemment à souligner l'enjeu de cohérence et d'exemplarité qui nous oblige sur ces travées. Il vise aussi, et c'est bien logique, à protéger ces établissements, puisque le virus entre aussi au

Monsieur le président, je vais vous donner l'avis de la commission, mais je sais déjà que le Premier questeur du Sénat souhaitera également prendre position sur ce sujet.

à un élu de la Nation l'accès à l'assemblée dans laquelle il siège. C'est une particularité qu'il faut tout de même entendre : nous représentons la Nation, avec les députés

avec le fonctionnement d'une assemblée constitutionnelle. Cela ne dispense pas nos assemblées d'adopter les règles nécessaires à cette exemplarité que vous avez revendiquée au profit de votre amendement, et que la commission des lois revendique

il n'y a pas de passe sanitaire, et il n'est pas question d'en instaurer un. S'il y a dans votre esprit l'idée qu'il y aurait un passe sanitaire pour l'accès aux lieux de travail en France,

de travail au Sénat, de risques sanitaires particuliers liés à la promiscuité, sauf à une promiscuité qui serait parfaitement volontaire et d'ordre privé. Nous n'allons donc pas établir privé. Nous n'allons donc pas établir spécifiquement pour nous des règles qui n'auraient pas de justification sanitaire et qui ne seraient appliquées nulle part ailleurs.

Nous souhaitons vivement, comme nous l'avons toujours fait au Sénat depuis le début de la crise sanitaire, que toute règle édictée pour nos concitoyens,

que, dans les conditions d'accès à la restauration collective au sein du Sénat, nous devrons transposer exactement les règles qui sont applicables au public. Nous le ferons,

d'un test récent assurant qu'ils ne sont pas contagieux. C'est toujours la même logique : ou bien nous mettons en place le passe sanitaire pour ces très grands centres, avec toutes les dérogations d'usage et une attention très importante portée au confort des consommateurs et à la capacité des Français à acheter ce dont ils ont besoin sans limitation ; ou bien nous nous exposons

Monsieur le ministre, vous connaissez l'exigence de notre commission en matière de sécurité sanitaire. Notre assemblée ne l'a d'ailleurs pas toujours suivie à cet égard. suivie à cet égard. Après beaucoup de débats et de réflexion, nous avons considéré, comme le Conseil d'État d'ailleurs, que la disposition envisagée par le Gouvernement était disproportionnée, par les contraintes qu'elle imposait par rapport aux objectifs sanitaires visés. Nous avons eu l'occasion d'en discuter ensemble, et vous m'avez expliqué qu'il existait de grands centres commerciaux comportant plusieurs grandes surfaces, dont certaines vendent du mobilier ou des équipements sportifs, mais aussi de grandes surfaces alimentaires ayant des activités multiples, avec des commerces, des restaurants, des pharmacies, des marchands de chaussures ou des bijoutiers : bref, c'est une ville dans la ville

vous n'êtes pas assujetti à la présentation du passe sanitaire. Mais si, dans cette rue piétonne, vous entrez dans des établissements où les risques de contamination sont spécifiquement élevés, vous devez le présenter. Il nous semble que l'on peut parfaitement transposer cette manière de faire aux grands complexes commerciaux. Il y aura, à l'intérieur du complexe commercial auquel le libre accès serait maintenu, des établissements pour lesquels il faudra un passe sanitaire et d'autres pour lesquels celui-ci ne sera pas nécessaire. Précisément, ces établissements pour lesquels il ne faudra pas de passe sanitaire ne doivent pas être interdits d'accès au public, parce que, à l'entrée du complexe commercial, celui-ci ne pourrait pas produire le passe sanitaire. Si nos concitoyens doivent faire leurs courses alimentaires de la semaine dans une grande surface alimentaire qui se trouve à l'intérieur du complexe commercial, il faut tout de même qu'ils puissent y accéder sans passe sanitaire, puisque, n'importe où où ailleurs, ils pourraient faire les mêmes approvisionnements sans passe sanitaire. Voilà pourquoi, monsieur le ministre, nous pensons que, sans porter préjudice à la sécurité sanitaire, les pouvoirs publics et les autorités sanitaires pourraient s'organiser autrement vis-à-vis des grands complexes commerciaux.

Cet amendement tend à préciser, en s'inspirant de la rédaction de l'alinéa 27 de l'article 5, que la réglementation objet de l'alinéa 14 de l'article 1 ne s'applique pas aux personnes n'accédant que pour l'exécution d'une tâche ponctuelle aux lieux, établissements, services ou événements soumis à condition d'accès pour motif sanitaire. Il s'agit, notamment, d'exonérer de l'obligation de présenter un justificatif vaccinal ou de dépistage les salariés des fournisseurs de ces sites, en particulier les chauffeurs-livreurs. Les personnels concernés interviennent en effet le plus souvent avant l'ouverture au public de l'établissement ou au tout début de l'ouverture, à un moment ou peu de clients sont présents, surtout dans la restauration.

On ne peut pas demander un passe sanitaire à l'entrée d'un bureau de vote ! Comme je vous vois venir, je le dis solennellement : on ne peut pas non plus imposer aux électeurs n'ayant pas de passe sanitaire de voter par voie électronique. N'y a-t-il pas déjà suffisamment d'abstentions dans notre pays, notamment chez les plus jeunes ? Mes chers collègues, vous savez comme la parole du Gouvernement peut être changeante ... Je vous propose donc de sacraliser l'expression démocratique essentielle, en interdisant définitivement, dès aujourd'hui, de demander la présentation d'un passe sanitaire à l'entrée d'un bureau de vote. Pas de passe sanitaire pour la démocratie

Votre intention est en fait de vous assurer que, l'année prochaine, ou à un autre moment, on ne dira pas aux électeurs : « Vous n'avez pas le droit d'entrer dans le bureau de vote

amendement est entièrement satisfait par le texte de la commission. Et je serais prêt à mener ce combat avec vous si certains voulaient remettre en cause cette exigence fondamentale de la démocratie.

n° 122 est-il maintenu ? Monsieur le président, j'ai écouté attentivement M. le rapporteur et M. le ministre : ils se sont adressés uniquement à notre collègue Hervé. Ils ne m'ont pas demandé de retirer mon amendement, donc je ne le retire pas

elle ne peut, pour l'instant, être aussi précise pour les enfants. » Ainsi, les conditions de sécurité ne sont pas réunies, nous semble-t-il, pour envisager la vaccination de la population des moins de 12 ans.

Je pense que, avant de faire la loi, il faut attendre que la science puisse nous éclairer. Interdire à l'avance les résultats d'une recherche clinique ne me semble pas conforme à la vision

Il est défavorable, monsieur le président.

de cette responsabilité ; d'autre part, c'est donner aux employeurs un accès aux informations médicales de leurs salariés. Je vous le rappelle, jusqu'à présent, les employeurs n'avaient pas le droit de posséder des informations médicales sur leur personnel,

Vous pouvez avoir un niveau élevé d'anticorps et une protection très faible, et, à l'inverse, des anticorps peu détectables, mais acquis d'une manière qui a conforté l'immunité et qui assure une bonne protection. Une sérologie ne permet donc pas de décréter que quelqu'un n'est pas à risque de développer la maladie,

Je le redis, aucune instance sanitaire ou scientifique ne va dans ce sens, et je ne prendrai pas la responsabilité d'autoriser la reconnaissance de vaccins dont je ne suis pas certain de la sécurité et de l'efficacité pour nos concitoyens.

aurons-nous protégés. Il n'y a pas deux catégories de Français en termes de protection sanitaire : ceux qui vivent à l'étranger, pour lesquels, tant pis, vaille que vaille, à la guerre comme à la guerre, et ceux qui vivent sur le territoire national et à qui l'on imposerait des exigences de sécurité pour leur santé.

prévu une dérogation au principe du secret médical, qu'elle a réservée aux professionnels de santé. Je pense, et vous me le confirmerez, monsieur le ministre, que le présent texte va au-delà,

on permettrait aux services de contrôle d'avoir accès à une donnée sensible pour aller dans certains pays étrangers qui en exigent la production, alors qu'on ne l'admet pas en France. La réponse est malheureusement assez simple.

Notre groupe s'oppose à la systématisation et à la généralisation du contrôle, qui doit demeurer exceptionnel et ne peut pas s'exercer sur une base quotidienne. Circonscrire les opérations de contrôle du passe aux officiers de police permet de les coupler directement aux opérations de contrôle d'identité, afin que le contrôle soit sensé et efficace. Par ailleurs, nous voulons exclure du contrôle toute personne non dépositaire de l'autorité publique, afin que ce contrôle demeure légitime et puisse s'effectuer en minimisant les heurts. Il s'agit de passer d'un contrôle systématique par chacun à un contrôle ponctuel et aléatoire effectué par les forces de l'ordre. Quel

Les dispositions relatives aux obligations imposées aux salariés ont incontestablement été améliorées par la commission des lois. toujours pas, en bout de course, une fois les procédures de conciliation épuisées et en l'absence de possibilités de reclassement, d'éviter une décision de licenciement. En conséquence, nous continuons de penser que le dispositif est excessif. Il nous paraît également inadapté, car il va produire des effets définitifs, alors que le cadre légal qui l'autorise est limité dans le temps, sa durée ayant même été réduite par la commission des lois.

Le présent amendement vise à supprimer la suspension du contrat de travail des employés de la restauration et du transport en cas de non-vaccination. telle disposition coercitive représente une discrimination en fonction de l'état de santé. Elle apparaît disproportionnée au regard des justifications sanitaires, de ses conséquences sociales négatives et de la désorganisation économique qu'elle risque de provoquer.

jamais les organisations syndicales de salariés. Pourtant, toutes sont favorables à la campagne de vaccination et à l'obligation vaccinale pour certaines professions.

? Inclure la restauration pénalise avant tout les travailleurs les plus précaires et les emplois saisonniers ou en contrat court. Ces emplois sont occupés par des populations elles-mêmes déjà fortement touchées par la crise,

a cinquante-quatre ans. Elle travaille depuis longtemps, et elle a continué de travailler tout en élevant ses deux enfants. Elle et son mari se sont toujours démenés pour que leur famille ne manque de rien.

mois. Elle fait quelques sacrifices pour les vacances de la famille. Elle collectionne les bons de réduction. Elle demande même de l'aide à des proches. C'est dur, mais elle se dit que cela finira par s'arranger et que, tant que l'on à manger et un toit, il y a plus malheureux. C'est aussi une femme de conviction, très attachée à sa liberté. Comme tous les Français, elle a accepté d'être enfermée pendant plusieurs mois, et elle n'était pas la dernière à se mettre à la fenêtre pour applaudir les soignants. Mais Véronique a un nouveau problème, auquel elle ne s'attendait pas. On lui a dit que, si elle voulait continuer à travailler, elle devait se vacciner. Sauf qu'elle ne veut pas- et c'est son droit le plus strict. Elle est donc confrontée à un choix cornélien. Comment continuer à travailler sans s'injecter ce vaccin, dont elle ne veut pas, alors qu'elle a un besoin vital de percevoir son salaire ? Avant de faire passer cette loi honteuse, je demande à chacun d'entre vous, ministres et sénateurs, de prendre cinq minutes de réflexion après vous être mis à la place de ces millions de Véronique qui se battent au quotidien pour leur famille. Prenez quelques instants et envisagez l'insupportable pression que vous leur faites subir, surtout si vous avez été privilégiés et que vous n'avez jamais passé des heures à faire les comptes le soir après le travail la perspective de perdre son boulot dans la période actuelle, simplement parce que l'on veut user, sans en abuser, de sa liberté ! Ces millions de Français tiennent ce pays à bout de bras. Ils ont tout accepté, parce que l'effort était collectif. Mais là, votre loi va permettre aux employeurs de les virer. même les soignants, passés en quelques mois du statut de héros de la Nation à quasi-criminels s'ils refusent de se faire piquer ! Aujourd'hui, 10 millions de Français survivent sous le seuil de pauvreté, et des centaines de milliers d'entreprises sont à l'agonie à cause de vos décisions politiques. D'autres ont perdu le fruit du travail de toute une vie. Et vous voulez faciliter le licenciement des travailleurs ! Ce n'est plus seulement une loi autoritaire et liberticide ; c'est une flétrissure pour toutes celles et tous ceux qui auront commis la faute de la voter

nos jeunes, qui se sont retrouvés en pleine incertitude sur leur avenir professionnel, à la fois démotivés face à une situation qu'ils ne contrôlaient pas et victimes d'une pandémie qui les touchait pourtant peu. Le Gouvernement n'a cessé de défendre leurs intérêts avec une ligne claire, que nous soutenons : accompagner tous les jeunes vers l'emploi. L'alternance a été l'une des mesures phares du plan « 1 jeune, 1 solution ». Son succès est indiscutable. La gestion de la crise ne doit pas risquer de dresser de nouvelles barrières à l'insertion des jeunes et d'aller à l'encontre de ce qui a été fait depuis plus d'un an pour les accompagner.

L'alternance est une chance pour l'avenir. Gérer la crise sanitaire est une nécessité pour tous. Nous pensons que les deux doivent être assurés. L'amendement

Un salarié qui serait suspendu se verrait convoqué à un entretien avec son employeur trois jours après son refus ou son incapacité à fournir un passe sanitaire, un certificat de rétablissement ou un test PCR négatif. Une telle disposition pose à nos yeux deux problèmes majeurs.

de leur situation médicale. Certes, la médecine du travail a pris ces dernières années beaucoup de coups et elle est particulièrement affaiblie. Une nouvelle fois, les salariés payent les décisions des gouvernements successifs, et pas seulement du vôtre.

que le Gouvernement daigne procéder à l'ensemble des consultations auxquelles il était tenu. Malheureusement, et comme le relève le Conseil d'État dans son avis, il faut faire avec cette absence de consultation. D'ailleurs, le Conseil d'État va encore plus loin, car il considère que ces dispositions ne peuvent pas être retenues faute de l'avis du Conseil commun de la fonction publique. Sur

généraux. Je m'interroge. Quelle procédure sera mise en oeuvre lors de la cessation de fonction ? La commission administrative paritaire sera-t-elle saisie ? Si oui, la non-présentation du passe sanitaire vaudra-t-elle faute disciplinaire ?

est donc totalement déconnectée de notre droit de la fonction publique. Or ses conséquences sont importantes et dramatiques pour les agents, dans des proportions qui dépassent largement le fait générateur. Si on pouvait éviter l'arbitraire, ce serait excellent

En effet, il s'agit d'une inquiétante dérive vers une société de contrôle, dans laquelle des citoyens auraient pour devoir de surveiller les autres, sous peine de se voir sanctionnés par les forces de l'ordre, qui vont donc se sanctionner elles-mêmes pour s'être contrôlées elles-mêmes ... On arrive tout de même à des situations rocambolesques

Le Syndicat national des espaces de loisirs, d'attractions et culturels évoque une baisse d'affluence potentielle d'au moins 70 % en raison du passe sanitaire, alors que les acteurs du secteur font tant d'efforts pour faire respecter les protocoles et surmonter les difficultés créées par des mois de fermeture imposée. Nous ne voulons pas de dystopie du type de ! Ce sont les professionnels et les Français, vaccinés ou non, qui refusent ce flicage de masse et cet État de plus en plus policier pour les honnêtes gens. Ce Léviathan administratif et liberticide vient gâcher les vacances d'été et le coeur de notre douce France, fondée sur le lien de voisinage et de fraternité. Chers collègues, ne faisons pas reposer le poids de ce passe autoritaire sur les épaules des professionnels. Ils ne sont pas des auxiliaires de police. Ils sont déjà asphyxiés de contraintes administratives et fiscales.

Cet amendement vise à supprimer le contrôle du passe sanitaire par les employeurs dans les entreprises et la sanction de fermeture administrative temporaire de leur établissement en cas de non-respect de ce contrôle. Notre groupe s'oppose à une société du contrôle généralisé. Le contrôle de la vaccination des employés et du passe sanitaire ne doit être effectué que par des personnes dépositaires de l'autorité publique ou par la médecine du travail, sous peine de porter un préjudice supplémentaire aux libertés publiques. Faire porter une responsabilité sur les employeurs est préjudiciable à la sérénité des relations de travail et risque de les dégrader inutilement. Les informations contenues dans le passe sanitaire doivent, le plus possible, demeurer confidentielles. n'ont pas à être portées à la connaissance de l'employeur, sous peine de porter atteinte au secret médical. La vaccination au sein des secteurs mentionnés au présent article doit au contraire être contrôlée de manière aléatoire par les forces de l'ordre.

a fait couler beaucoup d'encre : la pénalisation des sanctions pour les personnes soumises aux obligations de respect du passe sanitaire. Le Conseil d'État a permis que ces peines soient largement revues à la baisse par rapport à ce qui était prévu dans l'avant-projet de loi, en transformant ces sanctions en amendes de cinquième classe. Pour autant, en cas de récidive, l'article prévoit toujours une peine d'emprisonnement d'une année et une amende pouvant aller jusqu'à 9 000 euros.

Le régime d'obligation de présentation d'un passe sanitaire donne logiquement lieu à un régime de sanctions qui s'y attache et vient le rendre concrètement contraignant. Nous sommes opposés à l'ensemble de ce schéma, mais

lieux, établissements et événements concernés par l'application du passeport ou du passe sanitaire devront présenter à leur employeur ledit document pour pouvoir exercer leurs fonctions. Le projet de loi prévoit que les données contrôlées ne peuvent pas être conservées ou réutilisées à d'autres fins par les personnes ou services autorisés à contrôler les documents constituant le passe sanitaire. Par dérogation à ce principe, et sous réserve de l'accord du professionnel concerné, l'employeur peut conserver le justificatif de statut vaccinal du professionnel jusqu'au 31 décembre 2021. Cette disposition a pour objectif d'éviter aux professionnels vaccinés de présenter quotidiennement leur passe sanitaire à leur employeur. Afin d'assurer une mise en oeuvre efficace de cette dérogation, le présent amendement prévoit d'autoriser les employeurs à délivrer à chaque salarié l'ayant préalablement accepté de manière expresse un titre spécifique visible ou facilement présentable permettant de simplifier et d'accélérer la vérification de leur statut vaccinal.